Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c’est

Sénateur de l’Isère pendant dix ans, de 2001 à 2011, Louis Mermaz fut un témoin privilégié et un acteur de premier plan de la vie politique de la V République. Mes premiers mots iront à sa famille ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui ont partagé ses engagements et l’ont accompagné tout au long de sa vie, jusqu’à ses obsèques qui se sont déroulées le jeudi 22 août en l’église Saint Pierre de Limours et auxquelles j’étais moi même présent. Ce professeur agrégé d’histoire fut un fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand. Il écrivit dans ses mémoires : « J’avais été dès le début attiré par le rayonnement de François Mitterrand parce qu’il était porteur d’une ambition pour le pays. Avec lui, je savais que je contribuais à l’accomplissement de mes rêves. » Il est à ses côtés dès 1957 au sein de l’Union démocratique et socialiste de la Résistance

En 1971, après le congrès d’Épinay, il devient membre de la direction nationale du parti socialiste ; il y est chargé des fédérations. est ensuite au cœur des campagnes présidentielles de 1974 et de 1981. Après l’élection de François Mitterrand le 10 mai 1981 et les élections législatives qui s’ensuivent, il est élu président de l’Assemblée nationale. Il souhaite alors garantir le rôle du Parlement face à l’exécutif et lui rendre « ses droits et sa dignité ». Cet homme discret s’imposa comme une figure incontournable de l’État en alternant de hautes responsabilités à l’Assemblée nationale et des fonctions ministérielles dans les gouvernements de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, d’Édith Cresson et de Pierre Bérégovoy. En parallèle de son ascension politique au niveau national, Louis Mermaz cultiva son ancrage local en devenant maire de Vienne, mandat qu’il exerça pendant trente

En tant qu’élu local, Louis Mermaz n’eut de cesse de dénoncer, de la part de l’État, « une politique qui […] conduit de plus en plus à l’apparition de petits déserts administratifs

Il fut également membre de la commission d’enquête sur l’immigration clandestine, qui rendit ses travaux en 2006, et participa avec passion et opiniâtreté aux débats en séance sur tous les projets de loi relatifs à l’immigration, à l’intégration et au droit d’asile, sujets qui furent le point focal de son mandat sénatorial. Sa très grande culture politique fut précieuse à notre assemblée. Au delà de l’homme d’État, nous garderons dans nos mémoires le souvenir d’un homme affable, doté d’un esprit vif et d’un compas moral inébranlable.

Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie attristée et nos sincères condoléances à son épouse Annie et à sa fille Laure, ainsi qu’aux membres du groupe socialiste et à tous ceux qui ont partagé ses engagements

et un homme d’État, ce qu’il démontra dans ses différentes fonctions. Il avait beaucoup d’humour et beaucoup de rigueur, et il eut cette grande qualité qu’est la fidélité politique : comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, il fut l’un des tout premiers compagnons de François Mitterrand,

notre incompréhension, quand nous constatons que le Gouvernement soutient la décision de Sanofi de vendre sa filiale Opella, qui produit le Doliprane, la Lysopaïne ou le Maalox, à un fonds américain Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu garantir que le Gouvernement exigerait un certain nombre d’engagements économiques et que cette vente ne remettrait en question ni la production de Doliprane en France ni l’approvisionnement du marché français.

Comment ne pas se rappeler que, durant la crise du covid 19, nous manquions cruellement de Doliprane ? Et que dire de la perspective d’une introduction en bourse dans trois ans et des risques associés d’une offre publique d’achat (OPA) étrangère ? Quelles garanties pouvez vous nous apporter à long terme ? Ma question est donc double.

Parmi les garanties exigées, qui sont en cours de discussion, il y a le maintien de l’emploi, non pas sur quelques mois, mais bien sur la durée,… Comment ? … le maintien de l’empreinte industrielle, le maintien de la recherche et développement et, bien sûr, la localisation du siège

un an déjà que Gaza est enfermée dans une spirale de destruction et de mort. Voilà un an déjà que le monde a pris conscience du double standard qui gangrène notre discours et nos actions. Cette vérité cruelle heurte nos consciences, mais elle perdure, insidieuse, dans nos actes et nos choix politiques. Voilà un an déjà que, dans notre propre pays, la voix de celles et de ceux qui réclament l’application du droit international est non seulement ignorée, mais caricaturée et criminalisée. un an déjà que, dans cette région du monde où la diplomatie française avait autrefois un rôle prépondérant, notre voix a été réduite au silence. Discréditée, elle est désormais le reflet d’une politique qui a tourné le dos à la justice et au droit. À force de fermer les yeux sur les violations du droit international, nous assistons aujourd’hui à une escalade dangereuse, et Israël, dans une impunité totale, se permet d’attaquer délibérément les troupes de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), pourtant garantes de la paix, parmi lesquelles se trouvent des soldats français. Pour autant, je refuse de perdre l’espoir que notre pays puisse regagner la place qui lui revient sur la scène internationale, mais cet espoir ne pourra se concrétiser que si nous rétablissons le respect du droit humanitaire le plus élémentaire. Dans ce contexte, monsieur le ministre, la France a t elle la capacité et la volonté de défendre avec vigueur une solution humanitaire immédiate et efficace à Gaza ? Concrètement, quelles actions proposez

Si, comme la France, tous les pays du monde avaient immédiatement appelé à un cessez le feu, à l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire, à la libération inconditionnelle des otages ;

si, comme la France, tous les pays du monde avaient consenti à sanctionner les colons extrémistes et violents en Cisjordanie ; si, comme la France, tous les pays du monde consentaient aujourd’hui à soutenir financièrement l’Autorité palestinienne ; et si, comme la France, tous les pays du monde continuaient de plaider pour une solution à deux États, un État de Palestine vivant en paix et en sécurité aux côtés d’un État d’Israël, alors sans doute, monsieur le sénateur, n’en serions nous pas au point où nous en sommes. Vous Vous appelez le Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, à en faire plus, et vous êtes là dans votre rôle, celui de contrôler l’action du Gouvernement. Mais je veux vous inviter, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous joindre à nos efforts et à vous saisir

chers collègues

Ma question s’adresse à Mme la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Madame la ministre, pendant longtemps, le Sénat s’est senti très seul – très seul ! – lorsqu’il alertait, chaque automne, sur la dérive des comptes publics, notamment de ceux de la sécurité sociale. sociale. On nous regardait comme des Cassandre au moment de balayer, chaque année, en nouvelle lecture, les amendements de maîtrise des dépenses que le Sénat avait introduits. Mais c’était oublier que Cassandre avait raison et que c’est pour ne pas l’avoir écoutée que Troie a connu la ruine. Aujourd’hui, madame la ministre, le Gouvernement semble avoir pris la mesure de la situation budgétaire et des risques que la France courrait à l’ignorer plus longtemps. Vous avez pris l’opinion publique à témoin et proposez des mesures de redressement des comptes. C’est très vrai dans le projet

Mais, si des efforts sont nécessaires, pour ce qui est de la sécurité sociale notamment, ils ne sauraient constituer le seul horizon d’acteurs qui, pour beaucoup, ont le sentiment d’être déjà au bout de leurs possibilités, dans un système qui fonctionne mal. Je pense aux soignants, aux personnels des établissements de santé, à ceux des établissements médico sociaux, et à tant d’autres. Madame la ministre, si nous approuvons la démarche d’assainissement des comptes, que pouvez vous dire aux acteurs du monde social et aux assurés sociaux ? Comment les convaincre que maîtriser des comptes à la dérive est synonyme non pas d’abandon, mais d’engagement pour l’avenir ?

par exemple auprès des médecins généralistes, qui verront le tarif de leurs consultations passer à 30 euros, comme cela avait été négocié avec eux par l’assurance maladie. Nous respectons aussi les engagements du Ségur,

la ministre de l’éducation nationale, si nous ne pouvons qu’être à vos côtés lorsque vous saluez l’engagement des personnels de l’éducation sur le territoire hexagonal et dans les outre mer, nous ne pouvons oublier ceux de notre réseau d’enseignement français à l’étranger. Ces personnels, à l’heure où nous parlons, se trouvent en Ukraine, au Liban, en Israël, au Burkina Faso, en Iran et dans 135 autres pays. Ils servent la France et les enfants de nos compatriotes, de toutes conditions sociales, grâce aux bourses scolaires. Leur dévouement fait notre fierté autant que celui de leurs collègues en France. Ils portent eux aussi les valeurs de la République, souvent dans des contextes où leur vie et celle de leur famille peuvent être exposées. Les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, réunis cette semaine à Paris, nous l’ont une nouvelle Notre réseau scolaire international, qui compte 600 écoles, voit ses effectifs d’élèves augmenter dans le cadre de l’objectif « Cap 2030 » fixé par le Président de la République. Plus de deux tiers des enseignants du réseau relèvent du droit local ; nous ne pouvons donc nous priver de l’expertise des titulaires de l’éducation nationale, véritables piliers de ce système. En 2019, une note de service a fait évoluer les conditions de détachement : l’on est passé d’une tacite reconduction à des détachements limités à deux périodes de trois ans. Si cette réforme pouvait se justifier à l’époque, elle a perdu de sa pertinence au regard de la recrudescence des conflits géopolitiques, des restrictions de déplacement qui ont prévalu pendant la crise sanitaire et des problématiques liées aux visas, entre autres. Désormais, les enseignants sont de plus en plus réticents à postuler pour l’étranger. De plus, la contrepartie promise lors de cette réforme était la valorisation des acquis de l’expérience. Tenir cet engagement et mettre en place à cet effet un groupe de travail devient impératif.

Ce réseau d’enseignement unique au monde permet à la France de tisser des liens diplomatiques, économiques et culturels, grâce à ses milliers d’anciens élèves, étrangers et français, mais aussi grâce à ses personnels. Madame la ministre, y a t il meilleur moment qu’aujourd’hui pour témoigner à ces derniers notre attachement et notre soutien ?

à davantage de personnels titulaires – tel était le sens initial de la mesure de 2018, et je sais que vous y aviez été, à l’époque, très favorable. Je suis aussi consciente des difficultés de l’expatriation : je connais ses défis, et je connais aussi ses désillusions,

Je regrette cependant le retard pris dans la mise en place du groupe de travail que vous avez évoqué ; celui ci permettrait pourtant d’identifier les mesures pouvant être mises en œuvre avant, pendant et après le détachement. J’ai donc demandé que ce groupe de travail soit mobilisé au plus vite et que ses conclusions me soient remises à la fin de l’année 2024. Notre réseau, madame la sénatrice, est d’une qualité exceptionnelle, mais je suis aussi consciente des difficultés de recrutement que rencontrent certains de nos établissements. C’est pourquoi j’ai demandé une évaluation précise de chaque situation,

famille et de la petite enfance, mes chers collègues, en juin dernier, un arrêté, validant deux accords de branche, est venu étendre la « prime Ségur » à tous les salariés du secteur social, médico social et sanitaire associatif. Il s’agissait d’une demande ancienne de la part des acteurs du secteur, qui dénonçaient une injustice envers les « oubliés du Ségur », la prime ne visant à l’origine que certaines professions uniquement, notamment les soignants. Avec cet arrêté, les salariés ayant des fonctions administratives ou techniques en bénéficieront désormais. Cette extension de la prime sera financée par l’État, la sécurité sociale et les départements. Si l’on peut se réjouir pour les professionnels concernés, il n’en va pas de même pour les départements et les associations, dont la situation financière était déjà plus que fragile avant cet arrêté. Ils se retrouvent contraints par cette nouvelle mesure rétroactive, sans avoir été consultés au préalable. Les dotations insuffisantes, l’explosion du coût des matières premières, les revalorisations salariales, la hausse des prestations sociales qui leur incombent et l’effondrement des droits de mutation concourent à la dégradation des finances du département de Maine et Loire et, plus largement, de tous les départements. Beaucoup d’entre eux sont arrivés au bout de leurs capacités et ne pourront tout simplement pas financer la prime. Bientôt, il leur faudra choisir entre leurs missions, car il leur sera impossible de toutes les honorer. Les départements sont, avec les communes, l’échelon de proximité le plus direct pour les Français ; ils assurent un rôle particulièrement important dans les politiques sociales et de solidarité. Si l’on souhaite que les enfants et les personnes âgées ou en situation de handicap soient accompagnées dignement, que l’aménagement du territoire soit convenablement assuré ou que la culture continue d’être promue, il est nécessaire d’agir. Madame la ministre, êtes vous aujourd’hui en mesure de rassurer les départements quant à la compensation de cette nouvelle charge ? La parole

que je retrouve avec plaisir ! Madame la sénatrice Corinne Bourcier, vous mettez en lumière l’accord historique de revalorisation des professionnels du secteur sanitaire, social et médico social. Cet accord, qui a été conclu à l’unanimité, permet d’étendre la prime Ségur aux 110 000 professionnels qui n’en bénéficiaient pas jusqu’à présent. Surtout, il engage les partenaires sociaux de la branche dans une dynamique résolue de fusion de l’ensemble des conventions collectives existantes. Cette future convention collective unique mettra fin à une situation inadaptée où 20 % des salariés de la branche ne bénéficient pas de protection, où aucune garantie de progression des carrières en fonction des mouvements entre établissements n’est prévue aujourd’hui et où prédomine une grande faiblesse des rythmes d’évolution des salaires.

entre le Gouvernement et les départements, comme vous l’avez souligné. Une enveloppe de 500 millions d’euros a été dégagée, dont 120 millions pour les départements, qui a été revalorisée à 170 millions pour prendre en compte l’inflation. Comme vous le rappelez, plusieurs types d’établissements relèvent de la tarification et de la responsabilité des départements, que ce soit dans le secteur de la protection de l’enfance ou pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne la sécurité sociale, une enveloppe de 300 millions d’euros a déjà été dévolue à la branche autonomie pour l’année 2024. Des travaux ont été engagés engagés par les fédérations d’employeurs et présentés à la Commission nationale d’agrément avec les départements. Malheureusement, ces travaux ont été suspendus par la dissolution

La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

entre une ministre de la République et la porte parole du président directeur général du groupe EDF ?

de cette centrale que vous souhaitez m’interroger. Je vous répondrai très simplement. L’État est actionnaire d’EDF : il fixe le cahier des charges et EDF l’applique. Ce cahier des charges est connu : nous voulons pour Cordemais un projet industriel de reconversion qui soit durable et qui donne à chaque salarié de cette centrale un avenir. Cette centrale à charbon arrêtera sa production électrique en 2027. Elle sera la dernière à fermer

et qu’il correspond aux attentes des salariés. De plus, ce n’est peut être pas non plus le seul projet. En tout état de cause, vous pouvez compter sur moi pour l’investissement, ainsi que sur ma collègue Olga Givernet, qui suit de très près cette situation et travaille aux côtés d’EDF. La la ministre, une ministre de la République ne peut pas profiter d’un voyage en Loire Atlantique pour annoncer aux 350 salariés et à leur famille qu’ils vont perdre leur emploi, sans même prendre le soin de les rencontrer.

Enfin, une ministre de la République ne peut pas revenir sur la parole donnée. Pis, elle ne peut pas remettre en cause celle du chef de l’État qui s’est engagé en septembre 2023 centrale nous permettant d’aller vers la transition énergétique. C’est pourquoi, monsieur le Premier ministre, je m’adresse à vous. Comme vous, j’ai présidé un grand département. Nous savons l’un comme l’autre que la transition énergétique et la transition écologique ne se feront pas contre les territoires ni contre leurs habitants. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d’intervenir auprès du président directeur général d’EDF, M. Luc Rémont, pour lui rappeler simplement ses obligations et ses devoirs ! La parole est

et Républicain. Monsieur le ministre de l’économie, ce week end, dans une tribune, l’ensemble des parlementaires socialistes vous interpellaient pour que vous vous opposiez à la vente par le groupe Sanofi de sa filiale Opella, productrice du Doliprane, à un fonds d’investissement américain. J’étais moi même lundi matin sur le site de Lisieux, dans le département du Calvados, dont je suis élue, aux côtés des salariés pour vous dire de vive voix mon opposition ferme à cette vente. Personne n’a oublié que, en 2020, après la première vague de l’épidémie de covid 19, le Président de la République annonçait la relocalisation de la production de paracétamol en France avec un soutien massif de l’État. Quatre ans plus tard, nous apprenons avec stupeur la décision guidée par une logique purement financière de Sanofi, géant pharmaceutique français. Nous vous demandons solennellement d’empêcher cette vente, qui pose de sérieux enjeux de souveraineté sanitaire et constitue une menace directe pour les 1 700 emplois liés à l’activité industrielle et commerciale d’Opella en France. Comme l’a affirmé le Président de la République lui même, vous avez les instruments pour empêcher cette vente. Le décret Montebourg permet au Gouvernement d’opposer son veto au rachat de toute entreprise dont les activités sont essentielles pour garantir la protection de la santé publique des Français. Il faut l’utiliser et privilégier les alternatives françaises, au nom du patriotisme économique. Le Doliprane, médicament essentiel pour des millions de Français, ne doit pas changer de nationalité À ce propos, vous seriez bien inspiré de prendre connaissance du rapport du Sénat sur la reconstruction de la souveraineté économique de la France de notre collègue Franck Montaugé, ainsi que des travaux relatifs à la pénurie de médicaments auxquels a participé la sénatrice Émilienne Poumirol. Nous ne croyons pas aux possibles engagements qui seraient pris par Sanofi. Nous avons vu trop d’entreprises ne pas respecter leurs accords passés avec l’État, particulièrement en matière d’emploi, et préférer payer des amendes, même considérables. face à la crainte légitime d’une casse sociale à Lisieux, à Compiègne, et d’une délocalisation, dans un contexte marqué par des difficultés croissantes d’approvisionnement de médicaments, ma question est simple. Allez vous engager votre droit de veto ? Pourquoi ne l’avez vous toujours pas fait ?

de l’entreprise. Quel meilleur moyen de signaler l’importance que nous accordons à ce dossier ? Pour le reste, je le redis ici devant vous et je vous le garantis : rien n’est exclu et rien n’est interdit pour s’assurer de la production du Doliprane en France. La parole

Mais venez avec moi à Vitry, à Gentilly, ou à Montpellier : des centaines de postes sont déjà en voie d’être supprimés au moment où nous avons besoin de progrès contre le cancer ! À cela s’ajoute

dont le paracétamol. Où sont passées ces belles promesses de souveraineté ? L’État doit, monsieur le ministre, bloquer la prise de contrôle par une entreprise américaine. Sanofi doit respecter une mission d’intérêt

Si nous voulons avoir de l’emploi et de l’investissement en France – non pas uniquement dans le Doliprane et dans les génériques, mais aussi dans l’ensemble des technologies d’avenir –, si nous voulons vraiment que la France soit à la pointe de la recherche,…

publics et privés ? Croyez vous franchement que nous puissions envoyer le signal à l’ensemble des écosystèmes nationaux, européens et internationaux

examiner l’ensemble des dispositifs d’emploi qui sont en cours d’évolution dans notre pays. Vous avez raison, il s’agit là d’engagement, d’éthique, ainsi que de souveraineté industrielle et technologique. Pour le reste, sans me répéter, le maintien de l’emploi est la priorité absolue et ne sera pas négociable. Il ne s’agira pas de se contenter d’un accord en passant. Il ne s’agira pas de se contenter de mots. Nous aurons des accords formalisés – si le projet aboutit –, avec des garanties

nous nous engageons à ce que cette qualité d’accueil soit assurée dans tous les établissements de France. Il est important que les parents soient sécurisés. les parents soient sécurisés. Chaque matin, quand ils confient leur enfant à une crèche ou à une assistante maternelle, ils doivent pouvoir repartir l’esprit tranquille. Quand un enfant est confié à une structure de la petite enfance, il doit pouvoir y trouver les conditions de son épanouissement, de son éveil et de son développement. Je voudrais rendre hommage, ici, à tous les professionnels qui travaillent chaque jour dans ces structures de la petite enfance pour accompagner les enfants et améliorer les

Nous devons aussi nous assurer que les professionnels disposent des qualifications pour exercer leurs missions fondamentales. Nous devons également travailler à l’attractivité des métiers de la petite enfance, ce qui garantira l’épanouissement des enfants dans les structures d’accueil. nous devons, sous l’égide de la politique conduite par le Premier ministre, nous engager dans la voie du développement du service public de la petite enfance à partir de 2025 afin de définir

le cancer féminin le plus fréquent – 61 000 cas par an. Comme l’indiquent les rubans accrochés à nos vestes, le dépistage systématique permet de répondre à un enjeu majeur pour la santé des femmes. Si la campagne de sensibilisation est importante, encore faudrait il pouvoir accéder à ce dépistage. Les derniers chiffres de Santé publique France révèlent que moins d’une femme sur deux y participe. En cause, la faiblesse actuelle de notre offre de soins dans des territoires qui sont en voie d’extinction médicale. En Charente, département dont je suis élue, mais aussi ailleurs, les délais de rendez vous pour une mammographie excèdent souvent les six mois : ce n’est pas acceptable ! De surcroît, en Nouvelle Aquitaine, il est prévu une diminution de près de 30 % du budget alloué au centre de coordination des dépistages des cancers. On ne peut pas faire des économies aussi mal ciblées. En milieu rural, l’offre en radiologie n’est pas en mesure de faire face à la demande. Seules les capitales régionales ou Paris délivrent des rendez vous rapides pour celles qui, bien sûr, ont les moyens de se déplacer. Quand une femme a une ordonnance pour une mammographie, il faut impérativement établir le principe d’un rendez vous en urgence sous trois jours ce qui n’est vraiment pas le cas aujourd’hui. Madame la ministre, pouvez vous nous dire concrètement ce que vous entendez faire pour améliorer la prise en charge des dizaines de milliers de femmes confrontées à cette épreuve terrible du cancer du sein ?

Cavaillon a été le théâtre d’un acte de représailles d’une violence inouïe : quatre véhicules de police, dont trois sérigraphiés, ont été incendiés en plein cœur de ville, devant le commissariat. Cet acte criminel fait suite aux récentes opérations antidrogue, dites « place nette », menées avec détermination. Le message envoyé par ces criminels est clair : ils sont prêts à tout pour riposter. Notre réponse doit l’être tout autant : nous ne reculerons pas face à la menace. Ces représailles démontrent que les actions menées portent leurs fruits et touchent les réseaux criminels là où ça fait mal. Les dernières opérations ont conduit à vingt cinq interpellations. Par ailleurs, 6 kilos de cocaïne, 15 kilos de cannabis, 10 armes et 20 000 euros en argent liquide ont été saisis. Il est donc crucial, monsieur le ministre, de maintenir cette pression continue, implacable et déterminée. Je tiens à saluer

tous les moyens nécessaires. Monsieur le ministre, êtes vous prêt à renforcer, de manière pérenne, les effectifs de la police nationale à Cavaillon en accordant dix policiers supplémentaires et en réintégrant l’escadron de gendarmerie mobile déployé dans le cadre du plan national de sécurisation renforcée, qui nous avait été retiré pour les jeux Olympiques ? Êtes vous prêt, par ailleurs, à renforcer la brigade d’intervention d’Avignon qui est passée de dix neuf à neuf agents, et qui ne peut plus soutenir efficacement les circonscriptions de Cavaillon, de Carpentras et d’Orange ? Il est nécessaire d’y affecter au moins dix gardiens de la paix supplémentaires pour sécuriser les points de deal, éviter qu’ils ne se recréent dès le lendemain ailleurs et appuyer ainsi les opérations. Face à la violence et à l’impunité, seule une réponse forte, continue et résolue peut ramener la paix durablement à Cavaillon comme ailleurs. Dans cette guerre, votre soutien est essentiel.

Ensuite, les narcotrafiquants sont venus défier l’État. Ils ont riposté, brûlant quatre véhicules de police et allant jusqu’à endommager le commissariat. C’est absolument inacceptable ! Aussitôt, j’ai appelé le maire, Gérard Daudet, pour lui dire,

Nous ne nous sommes pas contentés de cela : nous avons mené, avec le ministère de la justice, une autre opération judiciaire, qui nous a permis de riposter, de porter de nouveau un coup et de procéder à de nouvelles interpellations. Voilà où nous en sommes. Vous avez, à juste titre, souligné la question des effectifs.

terrorisme. Nous n’avons pas gagné ce combat, qui est toujours à recommencer, mais nous avons porté des coups décisifs. Nous nous sommes totalement réorganisés. Ce que nous avons fait contre le terrorisme, il va falloir que nous le fassions

islamiste radical. Flambée d’antisémitisme, flambée des atteintes à la laïcité – on en compte 4 200 de plus depuis septembre 2023 –, multiplication des agressions d’enseignants,

Tous ces incidents ne sont pas dus au hasard : ils sont le résultat du grignotage de notre société par l’islam radical et par les Frères musulmans, dont nous finançons les associations directement ou par le biais de l’Union européenne. Je tiens la liste de ces financements à votre disposition – les deux minutes qui me sont allouées ne suffiront La Commission européenne vient de déléguer quatre programmes Erasmus à l’association Al Sharq, connue pour ses liens avec l’islam radical, et a intégré au programme la faculté des sciences islamiques de Skopje et l’université de Gaziantep, qui vient de rendre un hommage vibrant à Ismaël Haniyeh, ancien responsable du Hamas, avec – excusez du peu – 250 000 euros de subventions.

Je vais vous répondre de façon très précise, puisque vous avez cité le cas très révélateur de l’université de Gaziantep, au sud de la Turquie, qui a des liens très troubles avec l’islam radical et dont le recteur a rendu un hommage appuyé à M. Ismaël Haniyeh, tué dans une frappe israélienne après avoir commandité et dirigé le pogrom du 7 octobre 2023.

des affaires étrangères, chargé de l’Europe, une lettre à la Commission pour qu’elle se préoccupe de l’entrisme. Nous avons lutté contre le séparatisme. Il nous faut aussi, en France, sur le sol national, lutter contre l’entrisme. Je rends moi aussi hommage à ces deux professeurs,

La parole est à Mme Annick Petrus, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement a récemment évoqué une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion comme une piste pour percevoir des recettes supplémentaires. Cette mesure, confirmée par le ministre délégué chargé des transports, pourrait entraîner une hausse significative des prix des billets pour les liaisons entre les outre mer et la métropole, affectant particulièrement ces territoires. Dans un contexte où les populations ultramarines sont déjà lourdement impactées par le coût de la vie, cette augmentation risque d’accentuer la fracture territoriale et de peser encore plus sur les familles. Cette décision porterait également un coup grave à la continuité territoriale, essentielle pour maintenir le lien entre les outre mer et la métropole. Nous craignons également que cette décision ne provoque un effet de contagion des tensions sociales que connaît actuellement la Martinique, avec un risque de propagation des émeutes aux autres territoires, encore calmes. Les Saint Martinois, en raison de leur triple insularité, dépendent quasi exclusivement du transport aérien pour leurs déplacements et seront les plus durement touchés par cette nouvelle fiscalité. Monsieur le ministre, quand va t on enfin cesser de toujours prendre plus à ceux qui ont déjà le moins ? La parole

en particulier, de l’avion, non pas pour se déplacer, mais simplement pour vivre. La parole Nous serons attentifs, monsieur le ministre, car, pour nous, Ultramarins, la solidarité nationale signifie aussi le droit fondamental de pouvoir se déplacer à un coût raisonnable vers et depuis l’Hexagone. La continuité territoriale est un pilier essentiel de notre République, et il est inconcevable de pénaliser davantage des populations déjà durement touchées par le coût élevé de la vie, les contraintes liées à l’insularité et des revenus souvent bien inférieurs à ceux de la métropole.

chers collègues, nous sommes tous conscients de la situation de la justice en France. Le rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice a été publié aujourd’hui. Il confirme que la France se situe, malgré les efforts, en dessous de la médiane des pays du Conseil de l’Europe concernant les effectifs de la justice. Le coup d’arrêt à la programmation des crédits que porte le budget, c’est, concrètement, trois fois moins de postes de magistrats, de greffiers, d’agents pénitentiaires que ce que la trajectoire initialement prévue pour 2025 pouvait laisser espérer. Ce sont autant d’engagements et de promesses reniés Que dire aux professionnels du monde de la justice, confrontés, comme c’est le cas dans le département du Loiret, dont je suis élu, à des juridictions fortement sous dotées ? Que dire aux personnels des centres pénitentiaires, notamment au regard des engagements

à votre question et à votre soutien. Parfait ! Je suis persuadé que je le retrouverai lors de la discussion budgétaire… Complètement ! Vous avez voté une loi d’orientation et de programmation

! Aujourd’hui, notre justice est complètement engorgée à la suite d’une multiplication des dossiers dont elle est saisie. Nos concitoyens expriment leur attente

n’était pas acceptable au regard justement des engagements qui avaient été pris en termes d’effectifs et en termes de moyens. Je l’ai dit, le Premier ministre l’a reconnu, puisque le projet de loi de finances indique que ce budget fera l’objet d’un réajustement. Le Premier ministre s’y est engagé ; je lui fais, bien sûr, toute confiance.

Monsieur le président, ma question porte sur l’utilisation des caméras piétons. En 2019, face à l’aggravation des situations de tension et des actes de violence

Aussi, depuis le 1 octobre dernier, faute de texte, l’ensemble des agents de sécurité ne peuvent plus utiliser ces caméras piétons. Dès lors, je vous demande si le Gouvernement, qui a fait de la sécurité une priorité forte,

Vous pouvez aussi vous prévaloir de tous les agents de sécurité qui ont plébiscité ce dispositif, lequel a considérablement amélioré les relations

Votre ancien collègue Bruno Le Maire avait promis un texte pour la fin de l’année 2024, après un débat sur l’équilibre global du système énergétique, mais les événements politiques récents – je n’y reviens pas… – ont écarté cette solution peu convaincante. Je le rappelle, notre indépendance énergétique par le mix énergétique et la concrétisation des projets de développement hydroélectrique dépend de l’évolution du cadre juridique et de la résolution du contentieux européen sur le renouvellement des concessions.

Je connais ses lignes rouges, et j’y souscris : premièrement, pas de remise en concurrence ; deuxièmement, pas de mise en cause de l’intégrité d’EDF.

vous avez d’abord raison de souligner à quel point l’énergie hydraulique est une énergie adaptée à la situation : elle est pilotable ; elle est décarbonée ; elle est compétitive ; elle est durable. C’est une énergie dont nous pourrions augmenter les capacités si nous pouvions faire les investissements structurants que nous connaissons. Vous connaissez le sujet. Il n’est d’ailleurs pas nouveau, puisque cela fait quinze ans qu’un contentieux juridique nous empêche de mener à bien ces investissements avec la sécurité permettant aux concessionnaires de s’y engager. C’est d’ailleurs un sujet qui a résisté à de nombreux gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Comme vous l’avez dit devant la représentation nationale, la première solution serait évidemment une remise en concurrence.

En effet, l’industrie est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre en France et la chaleur représente 75 % de la consommation énergétique de l’industrie. Par ailleurs, la chaleur produite par fission nucléaire grâce aux prochains réacteurs modulaires offre une solution décarbonée et compétitive, qui permettra aux industriels de réduire fortement leur empreinte carbone. Cet amendement vise donc à étendre le champ des objectifs de la future loi quinquennale sur l’énergie en y intégrant explicitement la production de chaleur en plus de celle de l’électricité.

notre collègue Daniel Gremillet avait déjà proposé de faire adopter le principe de l’intégration de la construction des nouveaux réacteurs dans la loi quinquennale sur l’énergie. C’était l’article 4 de la loi.

du I de l’article L. 100 1 A du code de l’énergie dispose déjà que la loi quinquennale sur l’énergie fixe un objectif de développement des énergies renouvelables pour la chaleur,

de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution public d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article L. 2224 31 du code général des collectivités locales.

de ces trois amendements identiques ; pour les communes rurales ne disposant d’aucune solution de raccordement à un réseau d’électricité, de chaleur ou de gaz. Leur adoption ne me semble pas souhaitable : nous avons déjà inscrit un objectif en faveur des solutions pour les foyers ruraux non raccordés aux réseaux d’électricité, de gaz ou de chaleur au 2° de l’article L.

Le Gouvernement ne partage pas les motifs de cet amendement ; toutefois, les dispositions de l’article 13 apparaissent superflues dès lors que la programmation pluriannuelle de l’énergie a vocation à exposer la politique du Gouvernement dans tous les domaines de la politique énergétique et que les différentes synthèses et présentations qui en sont faites portent sur l’ensemble de ces

sécurité d’approvisionnement, défini à l’article L. 141 2 du code de l’énergie, ajouter les éléments d’information sur le coût global de cette source d’énergie ne relève en rien de la PPE, mais plutôt de rapports d’information distincts

Sur le fond, les données que vous demandez d’inclure dans la PPE sont largement publiques. Les investissements réalisés par EDF sur le parc nucléaire existant sont disponibles dans les documents d’enregistrement universel (URD) qu’elle publie. La mise à jour du rapport d’évaluation de 2022 sur le coût du programme de construction des six EPR2, porté

sont communicables. Le législateur et les différentes parties prenantes sont également éclairés par les rapports réguliers de la Cour des comptes. Ces rapports datant de 2005, 2014 et 2020 sont publics et comportent ces montants.

industrielles d’énergies renouvelables, parce que nos territoires ont besoin d’usines et d’emplois.

l’article L. 141 1 du code de l’énergie – à la Sfec. De la sorte, le Gouvernement devra exposer tous les cinq ans sa stratégie en matière d’énergie et de climat dans le cadre du document de synthèse accompagnant la PPE.

l’avis du Gouvernement ? La PPE est un plan dont l’existence a été introduite par la loi, tandis que la Sfec traduit la volonté du Gouvernement d’assurer une cohérence entre les différents exercices de programmation énergétique et climatique. Elle ne porte pas d’autre objectif que ceux qui sont traduits dans la PPE, dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et dans le plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc). Ce sont ces trois documents qui constituent, de fait, la stratégie française sur l’énergie et De plus, la loi prévoit déjà que la PPE permet de répondre aux objectifs de la loi de programmation relative à l’énergie et au climat. Cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait.

Nous ne souhaitons pas non plus que l’on revienne sur ladite loi, récemment adoptée, en élargissant la possibilité d’installer des SMR sans tenir compte du critère d’implantation à l’intérieur ou ou à proximité des installations nucléaires de base existantes. L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique, dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

l’avis de la commission ? Ces amendements visent à supprimer l’article 14, qui complète les souplesses administratives prévues pour la construction de réacteurs électronucléaires, dont les petits réacteurs modulaires, par la loi Nouveau Nucléaire du 22 juin 2023. ces amendements ne me paraît pas opportune. D’une part, l’article 14 n’a peut être pas fait l’objet d’une étude d’impact, mais il a profité d’un retour d’expérience dans le cadre du bilan annuel d’application des lois de notre commission pour l’année 2023 2024. L’ajustement ici proposé provient justement des acteurs de terrain. J’ajoute que la loi Nouveau Nucléaire, que l’article vient modifier, comportait une étude d’impact et avait fait l’objet d’un avis du Conseil d’État. D’autre part, l’article 14 ne pose aucune difficulté sur le plan de la sécurité et de la sûreté nucléaires. Les dispositions proposées ne s’appliqueront pas directement, mais nécessiteront un décret. Autre point : notre collègue Daniel Gremillet a déposé un texte dual, qui porte à la fois sur la programmation et sur la simplification énergétiques. Il est donc logique et souhaitable que ce texte pousse des mesures de simplification de ce type. Enfin, l’article 14 répond aux besoins des acteurs économiques. Je demande donc le retrait de ces amendements

Sortir de l’emprise des sites nucléaires existants ne correspond pas à l’équilibre voté en 2023. Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, que l’application de la procédure de droit commun pour les SMR est dans certains cas plus favorable que la procédure accélérée. Un travail de fond a été engagé avec les porteurs de projet de SMR. Il permet d’identifier si ces modifications législatives ou réglementaires sont nécessaires. Il pourra produire ses fruits dans quelques mois. Je vous invite à avoir une position de prudence d’ici là. La prolongation jusqu’en 2050 de l’application des mesures de simplification prévues par la loi d’accélération du programme nucléaire, ainsi que l’extension à cinquante ans de la durée maximale des concessions d’utilisation du domaine public maritime pour les projets de réacteurs liés à la résonance du nucléaire ne sont pas non plus nécessaires au développement de nouvelles installations.

en définissant un cadre spécifique pour des dispositifs expérimentaux implantés sur les sites de recherche nucléaires actuels, dans le strict respect des règles de protection de la population et de l’environnement ». Cette

Au contraire, nous souhaitons que la construction et l’implantation géographique des SMR soient avant tout conditionnées à l’élaboration d’une doctrine d’emploi de ces nouvelles technologies nucléaires.

les petits réacteurs modulaires dont la puissance thermique est supérieure à 30 mégawatts bénéficient d’un soutien public dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une qualification de projet d’intérêt général, et donc des souplesses administratives issues de la loi Nouveau Nucléaire.

Au cours du siècle à venir, la fréquence et l’intensité des catastrophes climatiques ne cesseront d’augmenter. Les inondations et submersions marines se multiplieront et le trait de côte reculera dans de nombreux territoires. Dans l’estuaire de la Gironde, il pourrait ainsi reculer de 479 mètres. En mars 2023, lors d’une audition au Sénat, Annie Podeur, présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, a souligné que les conséquences du changement climatique affectaient déjà, à des degrés divers, mais croissants, les réacteurs du parc actuel. Il est donc primordial pour notre sécurité collective de prendre en compte cette réalité. Nous ne pouvons déplacer les réacteurs existants, mais nous pouvons garantir la sécurité des futures installations. Monsieur Gremillet, vous estimiez d’ailleurs en janvier 2023 que cet amendement s’inscrivait dans la continuité de nos travaux, afin d’accélérer de façon responsable la production d’électricité nucléaire. Mes chers collègues, j’en appelle donc à votre bon sens et à votre cohérence.

n’a peut être pas fait l’objet d’une étude d’impact, mais il a fait l’objet d’un retour d’expérience dans le cadre du bilan annuel d’application des lois mené par la commission des affaires économiques pour l’année 2023 2024. D’autre part, l’article 15 ne pose aucune difficulté sur le plan de la sécurité et de la sûreté nucléaires.

Bien que le Gouvernement n’ait pas détecté de difficultés particulières relatives au cadre législatif applicable à cette installation très spécifique, nous restons ouverts au dialogue sur ce sujet. En tout état de cause, le Gouvernement réaffirme son soutien à ce projet international ambitieux,

trop lourdes, alors que ces sujets sont sensibles à l’échelon local. Il faut avancer très prudemment, car les compétences en matière d’urbanisme des communes ou de leurs groupements sont en jeu. Avec le dispositif proposé, le préfet aurait la main pour réaliser les mises en compatibilité nécessaires des documents d’urbanisme

monsieur le rapporteur,

Mon amendement a le même objet que celui que vient de défendre M. Jadot : cet article nous semble inutile, les intrusions de ce type étant déjà punies par des dispositions du code de la défense. En outre, le durcissement des peines semble disproportionné, puisqu’il ne repose sur aucune étude qui démontrerait les risques concrets de ces actions sur la sécurité nucléaire. En revanche, il est clair que cet article va dans le sens d’un renforcement de la criminalisation des militants et militantes pour le climat, approche que nous ne pouvons partager. La sécurité des installations nucléaires constitue certes un sujet majeur ; il convient qu’elle soit assurée

de telles infractions, c’est afin de renforcer la sécurité et la sûreté nucléaires. Par ailleurs, contrairement à ce qui figure dans l’objet de l’amendement n° 92, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré cette disposition sur le fond. Dans sa décision du 21 juin 2023 sur la loi Nouveau Nucléaire, le Conseil constitutionnel a simplement estimé que l’intégration de cette disposition à un texte à un texte relatif à la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires méconnaissait l’article 45 de la Constitution. Il s’agit d’un sujet de procédure, aucunement de fond. Je rappelle

320 000 tonnes de cet uranium appauvri, qui est simplement entreposé dans un certain nombre de hangars. À vrai dire, cet uranium appauvri représente un enjeu

! Quel est l’avis de la commission ?

pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée. L’uranium appauvri est déjà valorisé économiquement par la production de combustible MOX et n’a pas fait l’objet d’une qualification comme déchet, de sorte que son statut est aujourd’hui celui d’une matière.

des retombées fiscales existent déjà, la taxe sur les éoliennes maritimes et les cahiers des charges des appels d’offres. Le dispositif proposé à cet article créerait donc potentiellement un doublon. Quant aux projets de production d’hydrogène décarboné, ils ne génèrent pas

l’avis de la commission ? L’amendement du Gouvernement propose d’assouplir l’article 18, qui étend la contribution au partage territorial de la valeur aux projets d’éolien en mer et à ceux d’hydrogène renouvelable et bas carbone. Je suis très attaché à cet article, qui résulte des travaux

d’acteurs économiques et locaux. Pour autant, j’entends le besoin de souplesse et de gradualité dans cet élargissement du dispositif : d’une part, les projets d’éolien en mer sont spécifiquement assujettis à la taxe à la taxe sur les éoliennes maritimes ; d’autre part, les projets d’hydrogène renouvelable et bas carbone ne posent pas encore de fortes difficultés liées à des conflits d’usage. Dans ce contexte, je suis ouvert à ce que l’élargissement proposé soit facultatif, et non obligatoire : avis favorable.

M. Didier Mandelli. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Patrick Chaize, parlementaire que Mme la ministre connaît bien, puisqu’ils sont originaires du même département. L’objet de cet amendement est de résoudre une difficulté liée à la contribution d’urbanisme acquittée pour le raccordement des projets d’installations renouvelables au réseau de distribution d’électricité. Quel est article. Quel est l’avis de la commission ? a procédé à une réforme des réseaux de transport et de distribution d’électricité. Une partie de cette réforme a été réalisée par ordonnance, sur le fondement de l’article 26 de ladite loi. Toutefois, la rédaction retenue pour cet article par l’Assemblée nationale et le Gouvernement ne mentionnait plus le code de l’urbanisme dans le champ d’habilitation, de sorte

créé un traitement différencié entre les approvisionnements en électricité, d’une part, et en eau ou en gaz, d’autre part. Cette harmonisation rédactionnelle est de nature à favoriser la lisibilité du droit pour nos concitoyens et à limiter un éventuel risque contentieux. L’avis du Gouvernement

permet d’augmenter la puissance d’une telle installation sans modification du contrat de concession, lorsque les modifications impliquées sur ce dernier « ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135 1 du code de la commande publique

au sens de l’article L. 122 1 du code de l’environnement. Par ailleurs, l’autorité administrative peut autoriser temporairement une augmentation de puissance, sous réserve que le dossier de déclaration déjà mentionné ait bien été déposé, « en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national ». En effet, une telle augmentation de puissance se doit d’être encadrée. Il est bien précisé qu’elle ne doit s’appliquer que pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement » et qu’elle doit être proportionnée à la gravité de la menace en la matière.

Ces trois amendements identiques visent à supprimer l’article 20, qui facilite les dérogations aux débits réservés et les augmentations de puissance pour les installations hydroélectriques. Je ne suis pas favorable à une telle suppression. Tout d’abord, les dérogations proposées sont issues des travaux législatifs du Sénat. C’est notre

En tant que rapporteur, j’avais préféré opter pour la condition d’une « menace grave » plutôt que d’une simple menace, car le dispositif était nouveau, mais j’ai constaté, dans le cadre des travaux sur l’application des lois de la commission des affaires économiques pour 2023 2024, que l’existence d’une menace était suffisante. Plus encore, les dérogations proposées en matière d’installations hydrauliques sont suffisamment encadrées, car elles se contentent d’ouvrir une faculté pour l’autorité lui en faire une obligation, de sorte qu’une évaluation au cas par cas de l’existence d’une menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique et de l’opportunité d’une dérogation aux règles de continuité écologique est tout à fait possible. Enfin, les dérogations proposées

de l’autorisation. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne pour statuer sur l’avenir de l’hydroélectricité et relancer les investissements nécessaires. Le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation nécessiterait toutefois de modifier entièrement le régime de propriété des installations, par leur cession et la création d’un nouveau cadre juridique d’exploitation ; or la mise en place d’un tel régime ne peut se faire dans le cadre d’une expérimentation.

permet le passage à titre expérimental – j’insiste sur ce mot – des concessions hydroélectriques échues du régime des concessions vers celui des autorisations. Leur adoption n’est pas du tout souhaitable. Tout d’abord, notre commission et, je le crois, le Sénat dans son ensemble sont très attachés à l’expérimentation proposée, qui doit concourir à la résolution du contentieux européen gelant l’activité des concessions

Dans ce contexte, je souhaite que l’adoption de cet article 21 soit l’occasion, pour la représentation nationale, d’affirmer son soutien clair à une résolution rapide du contentieux pesant sur les concessions hydroélectriques. l’intérêt d’un éventuel passage du régime des concessions à celui des autorisations. C’est une faculté que nous ouvririons ainsi pour le Gouvernement. À charge pour lui de s’en saisir.

contraindre non seulement les installations de production d’électricité renouvelable raccordées au réseau public de transport d’électricité, mais également celles qui sont raccordées au réseau public de distribution d’électricité, à mettre à sa disposition leur puissance non utilisée aux fins d’équilibrage de l’offre et de la demande. Quel est l’avis de la commission ? amendement a un objet pertinent, puisqu’il vise à compléter le mécanisme d’ajustement, mentionné à l’article L. 321 13 du code de l’énergie, par lequel les puissances des installations de production d’électricité peuvent être mises à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE.

l’avis du Gouvernement ? L’exemption dont bénéficie le solaire photovoltaïque en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et d’artificialisation des sols est justifiée. Produisant de l’électricité injectée dans les réseaux, les installations photovoltaïques ont ainsi le caractère d’installations d’intérêt collectif et peuvent de ce fait être placées sur les terres agricoles et naturelles. Dans la très grande majorité des cas, les installations solaires thermiques produisent de la chaleur pour des usages privés liés aux processus industriels qui nécessitent de la chaleur, y compris l’été, surtout en cette Ces installations ne peuvent donc pas être implantées sur des espaces naturels agricoles et forestiers. Pour cette raison, il ne me paraît pas pertinent de leur appliquer le même régime d’exemption. Par ailleurs, les installations de stockage de ces énergies ne peuvent être comprises dans l’exemption, dans la mesure où les caractéristiques techniques de ces constructions artificialisent par nature les sols et ne permettent pas de de répondre aux critères de la loi de non atteinte durable aux fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Monsieur

et pas ailleurs, à savoir les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, mentionnées à l’article L. 141 5 3 du code de l’énergie, depuis l’article 15 de la loi du 10 mars 2023 relative en tant que rapporteur de ce texte, ai veillé à un équilibre entre accélération et contrainte, selon le souhait des élus locaux. D’autre part, il participe aussi d’une application du paquet européen Ajustement à l’objectif 55. Naturellement, l’encadrement ici proposé est sans incidence sur le sort réservé à la demande. C’est la raison

le cadre européen. Si l’article 16 de la directive RED III du 18 octobre 2023 prévoit bien que l’examen des projets d’énergies renouvelables doit être achevé dans un délai allant d’un mois à 45 jours, c’est seulement à partir du moment où l’administration dispose de suffisamment d’informations. le premier délai s’applique aux installations inférieures à 150 kilowatts ou aux rééquipements et le second délai aux autres installations. De telles conditions ne sont pas reprises dans l’amendement. D’autre part, s’il était adopté, cet amendement introduirait des complexités

puisqu’il tend à prévoir que l’examen de la complétude et de la régularisation du dossier doit être intégral. Pour la bonne instruction des dossiers, il est préférable que l’autorité administrative conserve la possibilité de demander des compléments durant toute la phase d’examen ; cela permet de sauver un grand nombre de projets EnR. EnR. La rigidité entraînerait sinon beaucoup de rejets de dossiers, incomplets ou irréguliers, une perte de temps pour tous, un renforcement des risques de contentieux, une obligation de redéposer des dossiers complets, donc une frustration pour les usagers. Enfin, la création de nouvelles décisions explicites et implicites liées à la recevabilité du dossier est également susceptible de nuire à la visibilité des procédures et de renforcer les contentieux sur les dossiers EnR. Par ailleurs, la réforme Industrie verte de la procédure d’autorisation environnementale, qui entre en vigueur le 22 octobre prochain, raccourcira de plusieurs mois l’instruction de ce type de dossier. Elle répond donc à vos préoccupations sur le fonds. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Gouvernement propose donc une approche qui conforte en particulier la CRE dans sa compétence à formuler des avis et ainsi son rôle potentiel dans les discussions européennes sur les sujets liés au marché de l’hydrogène.

Jean Jacques Michau. Le rôle de la Commission de régulation de l’énergie est de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz en France, au bénéfice de tous les consommateurs finals, que l’indique l’article L. 131 1 du code de l’énergie. Il s’agit d’une autorité de contrôle et de régulation des marchés de l’énergie. Cette structure n’a pas pour mission de concourir au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de et ce d’autant moins que ces technologies sont aujourd’hui controversées et que leur développement devrait faire en amont l’objet d’un débat démocratique. Ces technologies n’ont en effet à cette date fait preuve ni de leur fiabilité ni de leur efficacité et il n’est pas prouvé que le bilan carbone de l’utilisation de ces technologies soit vertueux. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas

Ils ne sont pas du tout opportuns. C’est la CRE qui a demandé que ces compétences lui soient attribuées dans ce domaine, dans le cadre de l’élaboration de la proposition de loi, puis à l’occasion des travaux de notre commission.

et de stockage du dioxyde de carbone. Reconnaître des compétences à la CRE dans ce domaine revient tout à la fois à accompagner, mais aussi à encadrer cette technologie : quoi de mieux qu’une autorité administrative indépendante

en cas de résiliation anticipée de contrats de fourniture d’énergie, notamment pour les petits consommateurs professionnels, génèrent de plus en plus de litiges. En effet, les petits professionnels ne bénéficient pas des protections du code de la consommation qui existent pour les particuliers, ces derniers pouvant changer de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel à tout moment. Les petits professionnels, eux, sont le plus souvent engagés auprès d’un fournisseur pour une durée déterminée, étant facturées en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture. Ces pénalités étant souvent d’un montant extrêmement élevé, elles les empêchent de résilier un contrat particulièrement désavantageux. C’est pourquoi, à l’instar du médiateur national de l’énergie, nous proposons que toutes les très petites entreprises soient exonérées des frais de résiliation anticipés, y compris en cas de contrat à prix fixe et à durée déterminée,

D’une part, elle n’est pas codifiée, de sorte que sa normativité interroge, de même que son articulation avec les autres dispositions du code de l’énergie ou du code de la consommation. D’autre part, elle n’est assortie d’aucune condition, ce qui signifie que son application serait nécessairement porteuse d’effets de bord, non seulement pour les fournisseurs, à commencer par le groupe EDF,

est à M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière de protection des consommateurs pour prévoir la publication d’un prix repère mensuel de vente du gaz naturel,

qui nous est proposé est pertinent. Il vise à appliquer des obligations prudentielles sous l’égide de la CRE. C’est une faculté ouverte par le cadre européen, en l’espèce le règlement du 26 juin 2024 sur l’organisation du marché de l’électricité. le Sénat a plaidé en ce sens, d’une part, dans une résolution adoptée le 1 juin 2023 sur l’initiative de nos collègues Daniel Gremillet et Claude Kern et, d’autre part,

Un rapport annuel ne semble pas nécessaire, dans la mesure où les modalités de la fermeture des centrales seront détaillées régulièrement par le Gouvernement et largement connues du grand public. Avis défavorable.

sont évidentes, nous devons rester humbles et ne nous fermer aucune porte. Ce qui doit guider notre action, c’est l’ambition d’avoir une énergie décarbonée et suffisamment pilotable. C’est uniquement ainsi que nous pourrons assurer notre sécurité d’approvisionnement et notre souveraineté énergétique.

au terme de cette discussion, il apparaît plus que jamais nécessaire que le Gouvernement dépose un projet de loi de programmation énergie climat dans le prolongement de la stratégie française pour l’énergie et le

un exemple, et pas des moindres : la taxation de l’électricité, voire du gaz, annoncée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour

Il vise à développer massivement, encore une fois sans tenir compte des coûts et des incertitudes, le nucléaire aux horizons 2040, 2045 et 2050.

l’objectif de 2020. Ne dites donc pas que nous respectons nos engagements européens ! Nous sommes montrés du doigt par la Commission européenne pour nos efforts insuffisants en matière d’efficacité énergétique. Et nous savons combien votre projet de budget va encore plus sacrifier les crédits en faveur du logement, dont nos concitoyens ont pourtant tellement besoin. Pour toutes ces raisons, nous ne soutiendrons pas ce texte. Nous espérons que le Sénat